Monsieur le président, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs les sénateurs, l'examen de ce projet de loi de finances rectificative en nouvelle lecture me donne l'occasion, au nom du Gouvernement,

Voilà encore quelques mois, monsieur le président de la commission des finances, vous plaidiez, aux côtés de M. le rapporteur général, pour obtenir un projet de loi de finances rectificative « limité aux seuls mouvements de crédits et mesures fiscales de l'année en cours ». Vous aviez raison, les collectifs budgétaires de fin d'année ont traditionnellement tenu le rôle de « voiture-balai servant d'exercice de rattrapage de la loi de finances, tant sur le plan fiscal que pour pallier les insuffisances de crédits du budget de l'année. Afin de répondre à ces dévoiements de la vocation initiale des lois de finances rectificatives, le Gouvernement a décidé de ne présenter aucune mesure fiscale, ni dans le corps du texte ni par voie d'amendements. De la même manière, le texte ne sera accompagné d'aucun décret d'avance : les ouvertures de crédits supplémentaires feront toutes l'objet d'un vote du Parlement, ce qui réhabilite le pouvoir des parlementaires. Permettez-moi de reprendre vos mots, monsieur le rapporteur général : « Nous ne pouvons que nous féliciter de ce que le PLFR de fin d'année retrouve son objectif d'origine, qui est bien de se concentrer sur les mesures ayant uniquement un impact sur l'année en cours. Nous comprenons d'autant moins la position de votre assemblée sur ce collectif budgétaire que celui-ci est aussi le point d'aboutissement de la démarche de sincérisation engagée par le Gouvernement depuis le début de la mandature. Vous avez vous-même salué cet effort la semaine dernière, monsieur le rapporteur général. Je vous cite de nouveau cite de nouveau : « Le projet de loi de finances rectificative que vous nous présentez correspond à une exécution plus saine des crédits que sous le précédent quinquennat ». De fait, ce texte suffit à démontrer la prudence des prévisions gouvernementales, ainsi que la sincérité des hypothèses retenues,

se borne quasi exclusivement à des annulations sur les crédits mis en réserve, à hauteur de 2,7 milliards d'euros, sans incidence sur aucune dépense opérationnelle des ministères. Il permet de faire face aux dépenses inéluctables de fin d'année, à hauteur de 2,1 milliards d'euros. Il permet de respecter les engagements pris dans le cadre du PLF pour 2019, qui fixait un objectif de dépenses de 600 millions d'euros en moins sur la norme de dépenses pilotables de l'État. Il n'y a eu cette année aucun surgel, aucune taxation interministérielle- le contraire du choix, puisque cette technique dilue les responsabilités -et nous avons, par ailleurs, dégelé plus de 2 milliards d'euros de crédits. Enfin, ce projet de loi de finances rectificative, à la demande de la commission du Sénat, sincérise » le schéma d'emploi des ministères. En rétablissant la sincérité des plafonds d'emplois, nous pourrons abandonner l'usage des schémas d'emplois. Nous redonnerons ainsi de l'autonomie aux gestionnaires publics, qui seront, dès lors, en capacité de piloter librement leur masse salariale, dans le respect des seuls plafonds d'emplois. sont, mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur le président, monsieur le rapporteur général, les raisons pour lesquelles le Gouvernement vous a fait part de son incompréhension face aux critiques portées à ce projet de loi de finances rectificative. En dépit En dépit de quelques divergences politiques, bien naturelles, je suis profondément convaincu que le changement de forme de ce collectif budgétaire de fin d'année est favorable à toutes et à tous, tant du point de vue de la portée de l'autorisation parlementaire qu'en raison de l'effort de sincérité engagé. La parole

Lors de l'examen de ce projet de budget rectificatif en première lecture, mon collègue Claude Raynal avait eu l'occasion de revenir sur le scénario macroéconomique, évoquant aussi bien les prévisions de croissance optimistes-

C'est peu dire que la politique de l'emploi est soumise, avec ce gouvernement, à une double peine. D'une part, les crédits de la mission connaissent une baisse drastique pour 2019. À périmètre constant, ils diminuent de 2,1 milliards d'euros en crédits de paiement.

territoires ultramarins et ruraux, l'accompagnement des enfants en situation de handicap en milieu scolaire et l'urgence sanitaire et sociale. Cela représentait, déjà, une diminution de 100 000 contrats aidés, avec, de surcroît, un taux moyen de prise en charge revu très nettement à la baisse.

Nous n'avions pas manqué de mettre en garde le Gouvernement contre les conséquences dramatiques de cette décision brutale, prise sans concertation et ayant entraîné, la fragilisation des petites associations et de certains services publics locaux, dans un contexte global de diminution des dépenses.

Dans les centres sociaux, ce sont 313 activités « petite enfance » qui ont été déstabilisées et 344 activités « jeunesse » qui se sont arrêtées. Depuis, le contrat

Comment justifier une telle sous-consommation, sinon en concluant que le Gouvernement a masqué l'importance de la baisse réelle du budget de ce programme ? Derrière ces crédits, combien, réellement,

l'appréhension des employeurs qui ne veulent plus recruter, car ils redoutent l'instabilité des annonces gouvernementales, et vous obtenez les raisons de la déconvenue organisée du PEC. Mes chers collègues, la réduction du nombre de contrats aidés est révélatrice d'une politique de l'emploi qui n'est malheureusement plus que la somme de variables budgétaires, au lieu d'être un vecteur réel d'amélioration de l'efficacité des parcours d'insertion. Les récents chiffres du chômage le prouvent

la même logique qui justifie que vous baissiez de 84,7 millions d'euros le montant de la subvention pour charges de service public versée à Pôle emploi en 2019. Cette anticipation, c'est de la politique fiction ! Car, malheureusement, les derniers chiffres du chômage sont mauvais,

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, nous examinons de nouveau le projet de loi de finances rectificative pour 2018, une semaine après la première lecture. Je crois que nous pouvons avoir un regret nos discussions se sont interrompues de façon prématurée lors de cette première lecture- c'est le moins que l'on puisse dire ! Malgré un avis plutôt positif de notre commission, alors que les premiers articles avaient été adoptés en séance, le Sénat n'a pas voté l'article d'équilibre.

En outre, il ne contient pas de mesure fiscale, ce qui doit être souligné. On pouvait donc légitimement penser que le Sénat allait, au moins, voter l'article d'équilibre. Cela n'a pas été le cas. Refuser la discussion est une posture qui affaiblit notre assemblée. Ça n'est pas satisfaisant ! Par principe, mon groupe estime que nous devons aller au bout de la discussion des textes,

subissons le retour de bâton de ce manque de dialogue. Et, évidemment, c'est un peu plus compliqué de résoudre les problèmes à froid que de les résoudre à chaud

nous étions plusieurs, dont Claude Raynal et le président Christian Cambon, à avoir déposé des amendements visant à rétablir cette solidarité interministérielle, en ligne avec l'article 4 de la loi de programmation militaire. Nous n'avons pas eu ce débat ; nous ne l'aurons manifestement pas non plus aujourd'hui. Il serait dommage que nous nous servions des discussions sur la mission « Défense » du PLF pour refaire le match. Nous devons faire preuve de cohérence et d'esprit de responsabilité. Sur la question de la transition énergétique, je partage les interrogations de nombreux collègues sur l'affectation de l'excédent de TICPE au budget général. Mais, encore une fois, nous n'en discuterons pas publiquement, alors que l'actualité commanderait un débat de fond, tel que celui que nous avons eu hier. Dans ce contexte, la commission mixte paritaire a bien entendu échoué et nous allons examiner une nouvelle motion tendant à opposer la question préalable.

il serait dommage que nos débats budgétaires n'aient plus lieu dans notre enceinte, mais se développent sur les réseaux sociaux. À force de dire que les débats au Sénat ne servent à rien, il ne faudrait pas que les Français finissent par le croire.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le groupe Union Centriste avait abordé l'examen de ce projet de loi de finances rectificative pour 2018

le secrétaire d'État, ce collectif budgétaire de fin d'année ne présente pas de dépenses fiscales et de mesures substantielles, se limitant à des ajustements de prévisions et de crédits. Le groupe Les Républicains le réclamait depuis des années ; il s'en félicite par conséquent. Cependant, ce projet de loi ne nous satisfait pas.

La réalité, c'est l'augmentation de la charge de la dette, avec 500 millions d'euros de plus que prévu, malgré la faiblesse des taux d'intérêt. Or 500 millions d'euros, c'est ce que coûterait le relèvement du plafond du quotient familial à son niveau antérieur, une mesure de rétablissement de pouvoir d'achat qui serait bienvenue pour les familles. Ce poids du service de la dette est la démonstration qu'il est nécessaire de diminuer notre endettement. La France se démarque, sur ce point, de ses partenaires européens. Les dernières données publiées par Eurostat font apparaître une baisse de l'endettement public au sein de l'Union européenne. Entre les seconds trimestres de 2017 et de 2018, l'endettement a ainsi diminué de 2,4 points dans toute l'Union européenne et de 2,9 points dans la zone euro. L'endettement moyen atteint 81 % du PIB des 28 États membres et s'élève à 86,3 % dans la zone euro. En France, la dette publique frôle désormais les 100 % du PIB. Après avoir atteint 97,6 % au premier trimestre de 2018, elle s'élève, au deuxième trimestre, à 99 % du PIB, selon les données publiées à la fin La dette de l'État, à elle seule, a progressé de 19,5 milliards d'euros sur le deuxième trimestre. Monsieur le secrétaire d'État, la réalité, c'est aussi que les dépenses en matière de transition énergétique ont été moins importantes que prévu en 2018, à l'instar de la part des taxes sur les carburants qui lui est affectée. La réalité, La réalité, c'est une diminution de 577 millions d'euros des crédits du compte d'affectation spéciale « Transition énergétique ». On ne peut pas reprocher à votre gouvernement de prendre en compte la décision de la Commission de régulation de l'énergie du 12 juillet dernier. Dans ce document très complet, on peut notamment lire que les volumes de production ont augmenté, en 2018, de 1,7 térawattheure, soit 3 % de plus que la prévision initiale, principalement du fait de la forte hausse de la production de l'énergie éolienne. Les énergies renouvelables poursuivent leur développement, ce dont nous pouvons nous réjouir collectivement. Si le coût public du soutien aux filières d'énergies vertes diminue, alors que les volumes produits augmentent, c'est tout simplement que les prix de marché ont augmenté. Monsieur le secrétaire d'État, le Gouvernement est piégé une nouvelle fois par la hausse des cours du pétrole. Toute politique de l'énergie doit nécessairement tenir compte de cet élément sous-jacent. Ce que nous reprochons à votre gouvernement, c'est d'affecter ces 577 millions d'euros de « cagnotte » au budget général. Eh oui ! L'augmentation, en 2018, des tarifs de la TICPE, taxe payée par l'ensemble des consommateurs d'électricité, ne sera malheureusement pas dédiée dans sa totalité aux actions en faveur de la transition énergétique. Vous renouvelez ici l'erreur de la trajectoire carbone. Comment rendre acceptables des taxes destinées à favoriser la transition écologique lorsque les recettes de ces dernières servent à financer tout autre chose ?

La réalité, c'est la fin de la solidarité interministérielle pour le financement des opérations extérieures qui prévalait depuis dix ans. Ce principe est pourtant inscrit à l'article 4 de la loi de programmation militaire votée en juillet 2018. Pour toutes ces raisons, monsieur le secrétaire d'État, notre groupe s'était abstenu en première lecture, ne pouvant cautionner la réalité de ces dépenses. D'autres groupes ayant voté contre le texte, celui-ci a été rejeté par le Sénat. La commission mixte paritaire ayant échoué, le groupe Les Républicains votera naturellement en faveur de la motion tendant à opposer la question préalable déposée par la commission des finances, dans la mesure où nos débats en nouvelle lecture ne pourront permettre de faire évoluer nos positions respectives. Nous pourrons ainsi reprendre plus rapidement nos travaux sur le projet de

Cette situation, qui n'a rien d'inédit, malgré les apparences, a évidemment de fortes chances de se reproduire aujourd'hui, et je dois dire que le dépôt d'une motion tendant à opposer la question préalable au texte issu des travaux du Palais-Bourbon participe à cette discorde constante. Permettez-moi cependant de trouver étonnant le traitement réservé à ce texte, dont la moindre qualité n'est pas la brièveté, loin des « voitures-balais » que nous avions pris la mauvaise habitude de traiter ces dernières années et qui produisaient bien souvent de mauvaises législations, sur lesquelles il fallait ensuite revenir. Notre surprise vient du fait que la loi de finances pour 2018 répondait à bien des objectifs auxquels la majorité du Sénat s'attache depuis longtemps ... Bravo ! ... suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune- vous pourriez m'applaudir, chers collègues ! -, progression générale d'une fiscalité alternative fondée sur la consommation, allégement de la fiscalité de l'épargne, avec la mise en place du prélèvement libératoire unique ... J'en passe. Nous sommes donc quelque peu surpris de la position de la majorité du Sénat. Se justifierait-elle par le fait que les dépenses publiques ne diminuent pas encore assez vite ? je vous invite, mes chers collègues, à une réflexion assez simple, venue au fil de nos débats de ces derniers jours, parce qu'il faut bien y voir l'une des sources du mouvement d'exaspération et de colère qui traverse le pays, de ronds-points en centres commerciaux, mais aussi les cortèges de retraités, de salariés et d'usagers de la SNCF ou encore dans les assemblées d'élus locaux : méfions-nous du sentiment de dégoût exprimé par certains devant l'usage qui est ou serait fait de leurs impôts, devant l'injustice qui préside en la matière. Ce qui renforce, en effet, la colère populaire, ce n'est rien d'autre que ce sentiment diffus qu'on ne sait plus faire le lien entre le fait de payer sa participation citoyenne aux charges publiques et les contreparties qu'on est en situation d'attendre ou de recevoir au terme de cet effort. Ce qui est, pour certains, une question de consentement à l'impôt, cet instrument nécessaire pour faire société et pouvoir vivre ensemble autrement que sous la loi du plus fort, est bel et bien : pourquoi cet effort Quand l'école publique perd une classe, quand la gare ferme, quand le bureau de poste réduit ses horaires d'ouverture, quand les services de l'équipement ne passent plus pour l'entretien des routes, quand la baisse des dotations aux collectivités les rend exsangues, la question vient naturellement. La question qui taraude

quelques chiffres, glanés dans l'évaluation des voies et moyens et les crédits de la mission « Remboursements et dégrèvements ». En 2018, nous aurons laissé pas moins de 98 milliards d'euros en allégements fiscaux destinés aux entreprises, plus 20,6 milliards d'euros plus 44,8 milliards d'euros de pertes de recettes sur l'impôt sur les sociétés, au titre de la « mécanique de l'impôt », plus les taux de TVA privilégiés, plus les exonérations de TICPE liées aux activités sectorielles à faible valeur ajoutée, plus les allégements et plafonnements de fiscalité locale, plus la ristourne dégressive sur les bas salaires. Il n'y a pas un impôt, une taxe, un droit quelconque pour lesquels on ne voie apparaître une exception, une dérogation ou un crédit d'impôt, dès lors que cela concerne les entreprises et particulièrement les actionnaires, et toujours au nom de l'emploi, de la compétitivité ou de je ne sais quelle baliverne, si l'on en juge par les chiffres du chômage et de la croissance. Je n'ai pas fait le total, mes chers collègues,

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, après l'examen avorté, et même frustrant, la semaine dernière, du présent projet de loi de finances rectificative, cette nouvelle lecture ne réserve pas de surprise, après un nouveau passage sans modification devant l'Assemblée nationale. Mes collègues ont déjà bien présenté les enjeux. Ce collectif de nature purement budgétaire, présenté le 7 novembre dernier, met à jour les prévisions macroéconomiques pour l'année 2018 et effectue des ajustements comptables, dans la perspective annoncée de « sincériser » le budget, pour reprendre le terme désormais consacré tant par les textes que par l'ambition gouvernementale. Je ne peux que redire ma satisfaction de ce retour à une pratique plus fidèle la fonction initiale du collectif budgétaire de fin d'année, malgré des délais toujours aussi contraints. Le déficit public est ramené à 2,6 % du PIB, contre 2,8 % en loi de programmation et en loi de finances initiale, ce qui traduit l'amélioration de la conjoncture constatée en 2017 et 2018. Le taux de dépense publique s'élève à 54,6 % du PIB, niveau proche de l'an dernier, mais en diminution. L'hypothèse de croissance est maintenue à 1,7 %, alors que l'INSEE se montre un peu moins optimiste, mais qui peut vraiment prévoir avec certitude son évolution ? Les erreurs de prévision des années passées, en négatif comme en positif, forcent, en la matière, à une grande modestie. La première partie du PLFR diminue de 38 millions d'euros les recettes du CAS relatif aux radars issues du produit des amendes forfaitaires et les réaffecte à l'Agence de financement des infrastructures de transport de La réaffectation au budget général de quelque 600 millions d'euros du compte d'affectation spéciale « Transition énergétique », qui a pu susciter des débats dans le contexte actuel, s'explique essentiellement par des raisons techniques, obligeant les comptes spéciaux à être en équilibre. le solde général est amélioré de plus de 5 milliards d'euros par rapport au projet de loi initial, bien que le déficit de l'État reste à un niveau toujours trop élevé, alors que les collectivités territoriales sont tenues, je le rappelle, à un strict équilibre budgétaire.

Je note d'ailleurs que, malgré l'amélioration, en exécution, du budget, on compte encore 300 millions d'euros de dépenses de personnel supplémentaires dans certains ministères. La tâche du Gouvernement

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues,

ces opérations sans qu'il soit nécessaire de recourir à la solidarité interministérielle et sans que cela remette en cause une seule commande de matériel, une seule dépense prévue au sein du ministère des armées. Nous

Je rappelle, en outre, que l'avis du Gouvernement est défavorable. En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit. Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Personne ne demande

Le scrutin est ouvert.

et sur Facebook. Au nom du Bureau du Sénat, j'appelle chacun de vous à observer au cours de nos échanges l'une des valeurs essentielles du Sénat : le respect des uns et des autres. Cela vaut pour les sénateurs comme pour les membres du Gouvernement et doit s'appliquer à l'intérieur comme à l'extérieur de cette enceinte. La parole est

Mais il y a quand même une vérité, et c'est la raison pour laquelle je m'adresse à Édouard Philippe. Votre majorité a été, ces derniers mois, ces dernières semaines, extraordinairement généreuse, généreuse de son mépris à l'égard de tous ceux et de toutes celles qui ne pensent pas comme elle. Ce fut d'abord, si vous me permettez de le rappeler, le hashtag #BalanceTonMaire. Ensuite, nous avons l'automobiliste, qui, nécessairement, fume des clopes », « roule en diesel ». Pourquoi pas des Gitanes maïs et pourquoi pas des « Pigeot mazout » ? Nous avons ensuite cette situation absolument invraisemblable des « gilets jaunes qui ont le mérite de tirer un signal d'alarme. Certes, ils le font à leur façon, qui n'est pas la nôtre, mais cela traduit sans doute un degré profond d'exaspération. Méritaient-ils d'être soupçonnés d'être manipulés par l'ultradroite et méritaient-ils, plus grave encore,

Plus tranquillement, je dirai que, plus grave que le mépris, il y a la pédagogie, qui est en fait votre condescendance à l'encontre des Français qui ne pensent pas comme vous. Il se trouve que l'on peut partager des opinions différentes : si les Français n'adhèrent pas à la loi de transition énergétique, c'est sans doute qu'elle est imparfaite. Ma question est très simple : allez-vous la changer

Le débat politique est vif, et il est vif dans tous les sens. Je pense que vous êtes, comme moi, attaché à la nuance et à la mesure. Il ne vous aura donc pas échappé, monsieur le sénateur, reconnaissons-le, que sur tous les bancs des deux assemblées, et parfois lorsqu'on est membre du Gouvernement, on subit des critiques, qui sont parfaitement fondées- c'est la démocratie et je ne m'en émeus en aucune façon -, qui sont parfois dures, dures, parfois peut-être un peu excessives. Elles sont même parfois blessantes. Chacun des ministres peut citer des exemples et chacun des parlementaires, dans sa vie politique, peut citer des exemples d'attaques

et je ne doute pas qu'un jour on me le reprochera, en faisant justement état d'une forme de condescendance. Il n'en est rien, j'essaie simplement d'utiliser les mots les plus adaptés et ceux que je crois les plus justes pour décrire une réalité qui est toujours complexe.

de la destruction de biens publics ou de violences, y compris à l'égard de forces publiques ? Le dire, monsieur le sénateur, ce n'est pas faire preuve de mépris, ce n'est pas faire preuve de condescendance : c'est simplement essayer de décrire une réalité qui, effectivement, est complexe, avec des mots que je crois justes. Vous m'interrogez- et c'est la deuxième partie de votre question -sur la perspective qu'a tracée le Président de la République, sur le cap qu'il a fixé en matière de transition écologique et notamment de trajectoire carbone. Le Président de la République a eu l'occasion de dire que ce cap avait été fixé, avait été présenté aux Français et qu'il n'en changerait pas. C'est un élément que je porte au débat ou, plus exactement, qu'il a porté ce matin au débat et que j'assume pour ma part parfaitement, devant l'Assemblée nationale comme devant le Sénat. Il a formulé toute une série de propositions tendant à ce que les mesures d'accompagnement que nous envisageons

nous allons le faire, oui, avec les associations de consommateurs ; nous allons le faire avec les élus locaux, qui eux aussi ont des responsabilités en la matière. Mais bien sûr, nous allons le faire avec les élus territoriaux, qui étaient d'ailleurs présents ce matin au Conseil national de la transition écologique. Nous allons le faire avec les ONG,

dans notre démocratie et dans notre République, c'est le Parlement qui fait la loi. Voyez-vous, monsieur le sénateur, dire cela, c'est exactement l'inverse du mépris, c'est exactement l'inverse de la condescendance : consulter les corps intermédiaires, nouer le débat avec les Français et ensuite en tirer les conséquences devant le Parlement, car c'est devant lui que les décisions se prennent. Quand je dis cela, monsieur le sénateur, je n'ai pas le sentiment de faire preuve de mépris ni de faire preuve de condescendance. J'entends des interjections, j'entends des « oh ! », je dis les choses telles que je les envisage en essayant de répondre de manière complète à votre question. La parole est à M.

Ma question s'adresse à M. le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, le Président de la République s'est exprimé ce matin. Sa parole était attendue. Du moins a-t-il mis du temps à aborder le fond du sujet qui traverse la société française : la question du prix du gazole et de l'essence. Mais c'est aujourd'hui chose faite. Le Président s'est exprimé à un moment où chacun mesure que la cohésion sociale est mise à mal. Le pays est au bord de la rupture civique. Je retiens de la parole présidentielle deux annonces pour parvenir à une transition écologique que nous souhaitons tous. Première annonce Mais est-ce bien là le dispositif que vous proposez ? Ou bien un dispositif ponctuel de baisse des taxes lorsque le prix du baril sera trop élevé ? Et là, je vous pose une question : pourquoi ne reprenez-vous pas simplement le dispositif que le Sénat a voté hier très largement, à savoir un moratoire, ce qui serait plus clair et plus net pour apaiser les tensions et préparer l'avenir ? Deuxième annonce du Président de la République : sa volonté de changer de méthode, volonté que vous venez d'illustrer à l'instant, monsieur le Premier ministre, et d'instaurer une écoute de nos compatriotes comme des corps intermédiaires. Vous le savez, l'effort fiscal est mal réparti, pour l'ensemble de nos compatriotes. En tout cas, ce sentiment est très largement répandu et c'est sans doute ce qui catalyse le malaise social. Ce malaise social est ancien, nous le savons tous,

qu'a eue le Gouvernement jusqu'ici de traiter un certain nombre de questions, peut-être avec une forme de verticalité. Comment souhaitez-vous et comment pensez-vous pouvoir demain restaurer la cohésion sociale ?

tout d'abord, je veux vous dire- je crois que M. le président du Sénat pourra en témoigner -que, pour ma part, je considère, dans cette période en particulier, qu'il faut faire preuve de la plus grande considération et du plus grand respect pour toutes et tous les élus, bien sûr, mais aussi les citoyens français, qui, parfois, se mobilisent et parfois expriment, dans la mesure où ils mettent de côté la violence, une forme de mécontentement ou de colère. Sur le fond de votre propos, vous le savez,

de ce que certains appellent la TIPP flottante, qui a été évoquée, là aussi, le Président de la République, le Premier ministre et moi-même avons eu l'occasion de dire qu'il fallait faire preuve de constance dans le temps

le Premier ministre vient de décrire notre démarche, qui est de construire des lieux de débat innovants sur les territoires, décentralisés, où pourront s'exprimer à la fois bien sûr les personnes qui sont actuellement mobilisées, ceux qu'on appelle les « gilets jaunes », mais aussi les élus locaux, les parlementaires, les associations, les représentants des syndicats, pour chercher ensemble des mesures complémentaires

Des milliers de manifestantes et de manifestants ont défilé samedi à Paris et dans toute la France pour faire entendre leur voix contre les violences faites aux femmes. Leur grande crainte était d'être invisibles, comme l'ont été pendant trop longtemps les violences sexistes et sexuelles. Toutefois, nous avons assisté à une mobilisation massive dans plus de cinquante villes en France. À l'appel du collectif « Nous Toutes ! » ont répondu près de 12 000 participants à Paris et plus de 18 000 dans toute la France. Nous devons évidemment saluer unanimement ce raz-de-marée violet qui touche la France dans son ensemble et qui manifeste une réelle révolte culturelle de la société, notamment contre les violences conjugales. L'étude nationale relative aux morts violentes au sein du couple a révélé ces chiffres : en 2017, 125 personnes dont 109 femmes, sont mortes victimes de la violence de leur partenaire. Déclarée grande cause du quinquennat par le Président de la République, l'égalité entre les femmes et les hommes est un enjeu majeur pour notre société et un combat culturel dont nous devons tous être acteur. Ce projet ambitieux est porteur de justice sociale dont chacune et chacun pourra bénéficier. Madame la secrétaire d'État, la réponse de l'État doit se faire à tous les niveaux.

Vous l'avez rappelé, il y a un an, le Président de la République a déclaré grande cause du quinquennat l'égalité entre les femmes et les hommes. À cette occasion, de nombreuses annonces ont été faites et plus de 127 mesures ont été lancées. Je ne les égrènerai pas toutes ici ; je citerai simplement quelques-unes d'entre elles, celles qui me semblent majeures. Nous nous étions engagés engagés à ce que le numéro d'appel 39 19 puisse répondre à 100 % des appels reçus : c'est fait ; à ouvrir dix unités de prise en charge des soins de psychotraumatologie pour les femmes victimes de violences : c'est fait- nous avons, avec la ministre des solidarités et de la santé, inauguré l'une d'entre elles cette semaine - ; à lancer une plateforme de signalement avec des policières et des policiers formés pour écouter les femmes et les hommes victimes de violences sexistes et sexuelles : cela a été fait ce matin avec le ministre de l'intérieur et la garde des sceaux. Nous avons fait voter également un certain nombre de dispositions, comme la transparence dans les écarts de salaire entre les femmes et les hommes, sur l'impulsion de la ministre du travail, Muriel Pénicaud. Nous avons mis en place les trois séances d'éducation à la vie affective et sexuelle, grâce au ministre de l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Nous avons lancé une grande campagne de sensibilisation pour mobiliser les témoins de ces violences sexistes et sexuelles, parce que nous avons besoin qu'ils agissent et signalent ces violences. Nous avons également fait voter- vous y avez pris part et je vous en remercie -l'allongement des délais de prescription pour les viols commis sur mineur et renforcé la formation des professionnels. Voilà un échantillon de ce que le Gouvernement a lancé en dix-huit C'est beaucoup, mais il reste encore un travail colossal à mener ensemble pour éradiquer les violences sexistes et sexuelles. Vous pouvez suivre les engagements du Gouvernement sur le site grande-cause-quinquennat.gouv.fr, et voir, ministère par ministère, où nous en sommes

Monsieur le Premier ministre, vous vous êtes rendu la semaine dernière au Congrès des maires et vous y avez défendu votre volonté d'un dialogue ouvert avec les édiles. Vous avez également salué leur engagement quotidien, exigeant et difficile. Des dispositions votées à l'unanimité par le Sénat correspondent à cet engagement. Nous sommes aussi amenés, en tant que sénatrices et sénateurs, à rencontrer les élus dans nos territoires, à dialoguer avec eux et à exprimer ici leurs préoccupations. Vous et moi connaissons leurs difficultés. Mais plus qu'être écoutés, les maires veulent surtout être entendus. C'est précisément ce que le Sénat, véritable creuset des voix de tous les territoires, s'attache à traduire dans ses débats, ses votes et ses délibérations. Car nous sommes avant tout des législateurs de plein exercice. Or les tensions qui agitent notre pays sont suffisamment préoccupantes pour que cessent les mesquineries qui ne font que décrédibiliser tous les élus. Mon groupe est convaincu que les collectivités locales, par leur proximité, ont un rôle prépondérant à jouer. Le Sénat de la République, lui aussi, avec sa légitimité, sa singularité et son expertise, doit être un acteur institutionnel de premier plan, aux côtés de l'Assemblée nationale, hors de tout corporatisme. Le prochain retour au Parlement de la révision constitutionnelle sera donc l'occasion de travailler à régénérer la confiance entre élus et citoyens. Nos élus locaux l'attendent. Mon groupe y travaille depuis longtemps. C'est dans cet esprit, monsieur le Premier ministre, que j'ai une proposition à vous faire, une proposition que le groupe du RDSE avait déjà portée ici en 2010 et qui reste d'actualité. Afin de renforcer les relations et le dialogue entre les élus locaux et l'État, êtes-vous prêt à avancer sur l'idée de donner le dernier mot au Sénat s'agissant, au sens de l'article 39 de la Constitution, des projets de loi relatifs à l'organisation des collectivités territoriales ?

j'ai été maire beaucoup plus longtemps que je n'ai été Premier ministre et il est absolument certain que cela ne changera pas.

parce qu'on a envie d'être debout et de participer à l'action publique. C'est un engagement admirable et vous ne m'entendrez jamais dire le contraire. J'ai indiqué que le Gouvernement était prêt à améliorer les conditions d'exercice du mandat. monsieur le président, par des considérations sur la fiscalité ; cela passe par la conciliation entre l'exercice d'une activité professionnelle et le mandat de maire, cela passe par des considérations sur la protection sociale, cela passe par un ensemble de considérations qui sont d'ailleurs assez différentes selon la taille des communes, selon les contraintes pratiques qui s'exercent sur les maires, selon l'assistance administrative dont ils peuvent disposer dans leur mairie.

non pas du statut de l'élu- je ne suis pas sûr que les élus veuillent un statut -, mais de l'amélioration effective des conditions d'exercice du mandat. J'ai eu l'occasion de dire à M. le président du Sénat la disponibilité du Gouvernement à cet égard. Nous allons travailler

Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, ce matin, le Président de la République a esquivé la question qui traverse les mobilisations, des « gilets jaunes » aux infirmières, des salariés en lutte pour l'emploi à ceux qui agissent pour les services publics dans l'Hexagone et outre-mer. Dans son discours de la méthode, il n'a pas répondu à cette question : comment concilier transition énergétique et justice sociale ? Il est resté silencieux sur ce que l'on entend partout : augmentez nos salaires, augmentez les pensions, aidez-nous à vivre, simplement à vivre ! Le Président a parlé d'une grogne, mais ce n'est pas une grogne ! C'est un ras-le-bol, une colère qui monte et dont vous ne mesurez visiblement pas l'ampleur et la diversité. La transition énergétique n'est pas en cause et le plaidoyer de M. Macron tombe à plat. Ce qui est en cause, c'est de la faire payer par les plus déshérités, par les classes moyennes. La question est : qui va payer la lutte contre ce changement climatique ? Notre peuple n'est pas stupide, il réfléchit ; il ne veut pas d'un accompagnement, il exige. Il voit bien que M. Macron ne bouge pas d'un iota sur sa politique de protection des riches. Ce dernier garde le cap, oui, mais le cap du CAC 40. Monsieur le Premier ministre, allez-vous enfin admettre que c'est ce « capitalisme cannibale » dénoncé par Nicolas Hulot qui détruit la planète ? Allez-vous contraindre les plus riches, ces actionnaires qui font primer leurs intérêts sur l'intérêt général et écologique ? fortune, l'ISF, annuler l'augmentation des taxes sur le carburant, augmenter dès le 1 janvier 2019 le SMIC de 200 euros : c'est une urgence sociale qui ne peut se satisfaire de promesses. Voilà ce que veut le peuple, qui a besoin non pas d'aumône, mais d'un changement maintenant. Allez-vous y répondre, monsieur le Premier ministre ? Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, madame la présidente Assassi, vous m'interrogez sur la question de la transition écologique et du pouvoir d'achat et vous nous indiquez ne pas avoir été convaincue par les propos tenus par M. le Président de la République ce matin. J'aurais aimé que vous le soyez ; je ne suis pas surpris que vous ne le soyez pas. Je voudrais essayer de répondre à la question que vous formulez en indiquant d'abord quelques éléments

solide. Le pouvoir d'achat, vous le savez, madame la présidente, a baissé de façon continue de 2008 à 2016. C'est un fait, je ne m'en réjouis pas, vous non plus, personne sans doute ici, mais enfin disons les choses : cette diminution du pouvoir d'achat a été importante au cours des dix dernières années. Les mêmes indiquent que, avec la politique du Gouvernement, il y aura, en 2018 et en 2019, une augmentation du pouvoir d'achat. Je tiens à le souligner et, en disant cela, je ne nie pas une seconde, madame la présidente Assassi, que ceux qui enfilent des gilets jaunes

Notre objectif, et c'est la différence entre nous, madame la présidente Assassi, n'est pas de répondre à cette interrogation en disant partout de façon indéterminée que le SMIC va augmenter de 200 euros- j'avais bien compris que votre proposition n'était pas de fixer le SMIC à 200 euros, mais bien de l'augmenter de 200 euros. Je comprends que vous formuliez cette proposition, car elle est conforme à ce que propose votre famille politique depuis très longtemps. Non seulement je n'y crois pas, mais je sais quel a été l'impact régulier des augmentations que vous décrivez, lorsqu'elles sont intervenues, sur le chômage, notamment sur celui des salariés les moins formés.

par le travail, par la diminution du chômage, par l'investissement, par l'attractivité du pays et en substituant à une fiscalité qui reposait sur le travail une fiscalité qui repose sur la pollution.

à la moyenne de la croissance européenne, au cours du dernier trimestre, et il en sera probablement de même cours du trimestre suivant- je l'espère en tout cas -, la croissance française est passée très au-dessus de la moyenne de la croissance européenne. Nous sommes en train de créer des emplois, nous sommes en train de favoriser les investissements étrangers, nous sommes en train de faire le pari de développer cette stratégie d'une croissance économique qui permet la création de richesses, puis sa redistribution. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour le groupe socialiste et républicain.

Ce matin, dans une intervention très attendue, le Président de la République a annoncé une série de mesures, notamment son souhait d'adapter la fiscalité du carburant au cours du pétrole. Ça tombe bien, monsieur le ministre, un amendement du groupe socialiste a été préparé en ce sens. Seulement, hier, en votre absence, votre collègue de Bercy a émis un avis défavorable sur cet amendement demandant l'instauration d'une TICPE flottante et présenté par notre collègue Roland Courteau. Nous sommes bien sûr heureux que nos arguments aient infusé dans la nuit pour convaincre le Président de la République. Toutefois, si cette TICPE répond à une partie de la colère actuelle, elle ne répond pas à la question fondamentale qui doit financer la transition écologique et sur quelles bases doit s'asseoir ce financement ? Sur l'ensemble des Français les taxes carbone ou la TVA, qu'ils soient riches ou pauvres ? Ou en faisant contribuer, comme nous le proposons, ceux qui en ont davantage les moyens, en rétablissant l'ISF ou en augmentant la que vous avez abaissée à 30 La majorité des manifestants, dont beaucoup habitent des territoires ruraux comme le mien, sont confrontés à une baisse significative de leur pouvoir d'achat et à des inégalités territoriales croissantes. Ils demandent plus de justice fiscale et sociale, et je ne suis pas sûr que les mesures annoncées y répondent.

Monsieur le sénateur, je vous présente mes excuses, si, par avance, vous pensez que, par mon attitude, je vous manque ou je manque au Sénat, mais il se trouve que j'ai passé, et j'en suis très heureux,

Sur le fond, je ne voudrais pas ne pas vous répondre, monsieur le sénateur Claude Bérit-Débat. C'est à bon droit que le ministère de l'action et des comptes publics, par l'intermédiaire d'Olivier Dussopt, vous a répondu défavorablement, parce que votre proposition, si elle est évidemment à étudier, n'est pas la même

Vous ne m'avez pas du tout convaincu, monsieur le ministre, et de plus, vous n'avez pas vraiment répondu à ma question. La TICPE flottante est exactement identique à ce que propose le Président de

Cette incompréhension se renforce lorsque les faits ne semblent pas correspondre aux propos. La question des méthodes de calcul des dotations aux collectivités locales est un sujet extrêmement important pour lequel des réponses précises sont attendues par nos élus. Le Gouvernement ne cesse de rappeler qu'il a stoppé la baisse des dotations engagée les années précédentes. Nous entendons ces propos, mais, dans les faits, nous sommes sans cesse alertés par nos élus qui voient leurs dotations baisser sans pouvoir obtenir d'explications des préfets ou de Bercy on parle d'une baisse annuelle de 10 % à 30 % des budgets pour certaines communes. Depuis des mois, de nombreux courriers ont été adressés à Bercy et aux préfectures pour obtenir des informations précises quant aux critères retenus et aux méthodes de calcul adoptées. Personne à ce jour n'a obtenu de réponse ! Dès lors, comment voulez-vous que les relations s'améliorent ? Comment voulez-vous que cessent cette exaspération et cette colère des élus locaux ? Lorsque les maires écrivent au préfet, on les renvoie à Bercy. Lorsqu'ils écrivent à Bercy, on les renvoie au préfet, car Bercy ne peut ou ne veut pas fournir de réponse. Et maintenant on les renvoie au ministère de la cohésion Tout le monde se renvoie la balle : ce ping-pong ne peut plus durer ! Monsieur le ministre, compte tenu des variations concernant les dotations, nous demandons au Gouvernement un engagement ferme pour répondre en moins d'un mois à chaque courrier de chaque élu local et lui fournir des explications détaillées sur les méthodes de calcul de ses dotations et les critères employés, en toute transparence. Au nom des élus locaux, pouvons-nous obtenir, monsieur le ministre, cet engagement ferme du Gouvernement ?

cette question, je me la suis posée moi-même lorsque j'étais maire de ma commune : les règles de calcul de la DGF ne sont pas évidentes, et cela ne date pas d'hier. Il est vrai que les variations sont parfois importantes

les grandes déstabilisations de cette année et de l'année dernière- c'est bien sûr la modification du périmètre des intercommunalités qui a conduit à revoir beaucoup de calculs en la matière. Votre question est précise, comment peut-on agir pour améliorer les choses ? Premier engagement : je vous propose de ne retenir qu'une seule adresse, celle de Jacqueline Gourault et la mienne au ministère de la cohésion des territoires. Le deuxième engagement

Qui dit stabilité veut donc dire aussi, peut-être, une DGF moins dynamique ; et si celle-ci est moins dynamique, cela veut dire aussi qu'on répond moins aux inégalités territoriales. C'est un beau débat Politique, avec un grand « plus de dynamisme, cela veut donc dire moins de stabilité, et plus de stabilité, moins de dynamisme. On en parlera dès demain avec la délégation aux collectivités territoriales du Sénat, puisque le président Bockel m'y a invité. La parole

Monsieur le président, mes chers collègues, ma question s'adresse à M. le Premier ministre. Je voudrais revenir sur un incident ayant eu lieu à la fin de la semaine dernière au Sénat- plus exactement à l'extérieur du Sénat au lendemain de la fin du Congrès des maires -, et qui nous semble grave pour le respect de nos institutions. Après avoir écouté les discours, nos élus locaux ont dressé un bilan implacable : le compte n'y est pas ! Les maires ont l'habitude d'agir quotidiennement sur le terrain, pendant que le Président de la République gesticule solennellement depuis l'Élysée. Quand le Sénat travaille à mettre de l'huile dans les rouages de la République, le Gouvernement répond par des déclarations et des tweets, jetant de l'huile sur le feu par des raccourcis malvenus. Après le rapport de Mathieu Darnaud et de Jean-Marie Bockel, notre amendement d'ouverture en faveur des maires des petites communes cherchait à réparer à une injustice passée, sans cynisme ni populisme ; juste de la justice Monsieur le Premier ministre, la situation du pays est fragile, la crise démocratique couve, les menaces populistes sont aussi présentes en France. Votre silence après le tweet malheureux du ministre des comptes publics vendredi et des déclarations incongrues du porte-parole du Gouvernement ce matin, méritait une réponse de soutien aux élus de la République et au fonctionnement de notre démocratie. Alors, monsieur le Premier ministre, quelles mesures allez-vous prendre aujourd'hui- aujourd'hui et pas demain -pour nos fantassins de la République que sont les maires de France ? Quelles consignes allez-vous donner à votre gouvernement afin qu'il respecte la République ? La parole

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, M. le Premier ministre m'a autorisé à vous répondre, monsieur Bascher, puisque je pense être légèrement concerné par votre question. Il y a le fond et il y a la forme. Permettez-moi d'abord de revenir sur ce qui est sans doute le plus important, en tout cas quand on aime la littérature : le style. Est-ce que, pour ma part, j'aurais dû être au Sénat vendredi ?

Je le dis bien volontiers,

Gouvernement -, lire les très nombreux tweets d'attaques personnelles auxquels j'ai eu droit, non pas avant-hier, mais depuis un an et demi. Je ne l'ai pas fait, parce que, vous avez raison, il faut élever le débat. Sur le fond, monsieur le sénateur, y a-t-il un problème de rémunération, notamment de fiscalité depuis 2007, concernant les élus des petites communes- et non pas des « petits élus » comme j'ai pu le lire ici ou là ? La réponse est oui.

Lors de la seconde délibération que le Sénat va demander, le Gouvernement sera-t-il favorable au fait de rétrécir, comme l'a demandé M. le Premier ministre, l'incitation fiscale des 1 500 euros d'abattement, jusqu'à 18 000 euros ? La réponse est oui, pour les communes les plus petites. Mais il ne nous paraissait pas raisonnable, reconnaissez-le avec moi, que les présidents de région, les présidents de département et les maires de grandes villes, dont j'ai été, bénéficient des mêmes avantages fiscaux que les maires des communes les plus petites. Il y va de l'égalité républicaine. M. Jérôme Bascher, pour la réplique. Monsieur le ministre, nous ne voulons plus de double discours ni de double langage. Les Français parlent un langage clair, eux ; ils ont raison, et les élus attendent, aujourd'hui

Monsieur le président, mesdames, messieurs les membres du Gouvernement, mes chers collègues, ma question s'adresse à M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. le 5 avril dernier, je vous interrogeais dans cet hémicycle sur les conséquences financières pour nos communes du prochain abaissement de l'âge de la scolarité obligatoire à trois En effet, depuis 1959, les communes sont tenues de participer, sous la forme d'un forfait, au fonctionnement matériel des écoles sous contrat d'association avec l'État. En abaissant l'âge de la scolarité obligatoire de six ans à trois ans, vous allez étendre l'obligation faite à nos communes. Cette évolution sera tout sauf symbolique pour celles-ci. Chacun d'entre nous connaît les coûts relatifs à la scolarisation d'un enfant en école maternelle, qui sont particulièrement importants. Il ressort de l'avant-projet de loi pour une école de la confiance » que « seules les augmentations de dépenses qui résultent de l'extension de l'instruction obligatoire sont de nature à ouvrir un droit à accompagnement Comprenez : si une commune finançait déjà sur la base du volontariat, pas d'accompagnement de l'État ; si une commune ne finançait pas, accompagnement de l'État. Monsieur le ministre, au sein de notre Haute Assemblée, il est un principe qui nous est cher : qui décide, paie. Si l'État décide d'abaisser l'âge de la scolarité obligatoire, et qu'il crée, de ce fait, de nouvelles charges obligatoires pour nos communes, il est tenu d'apporter une compensation financière à celles-ci, et à l'ensemble de celles-ci. Son raisonnement ne saurait se fonder sur « qui faisait quoi avant Monsieur le ministre, le groupe du RDSE a salué la décision d'abaisser l'âge de la scolarité obligatoire. Toutefois, cette décision engage nos communes. Le Gouvernement envisage-t-il bien de ne soutenir que les communes qui ne participaient pas

D'ailleurs, je salue votre intérêt pour l'école maternelle, qui n'est jamais démenti. Je souligne aussi le fait que votre groupe avait déposé une proposition de loi dans ce sens en 2011. Bien entendu, aucun des gouvernements précédents n'a suivi votre bonne proposition

L'instruction obligatoire à trois ans, vous avez raison, madame la sénatrice, va créer une obligation nouvelle pour les communes, je le reconnais bien volontiers. Donc, conformément à la Constitution, nous allons respecter ce qu'elle demande, c'est-à-dire compenser ces dépenses nouvelles. Vous avez rappelé la logique vers laquelle nous sommes en train de nous orienter, c'est-à-dire le fait de compenser les dépenses nouvelles, autrement dit des dépenses qui n'existent pas aujourd'hui. Nous avons évidemment travaillé sur ce point, en lien

de la Constitution, c'est-à-dire la compensation des frais supplémentaires ou, pour le dire plus clairement, de ce qui n'est pas dépensé aujourd'hui et que nous mesurerons, c'est-à-dire la différence entre les dépenses de l'année 2018-2019 et les dépenses de l'année 2019-2020. C'est un principe simple, clair et tout le monde peut le comprendre. La parole

Un an et demi après l'avènement du « nouveau monde », les Français sont désespérés, exaspérés ! Bien sûr, vous héritez d'un passif lourd, mais 73 % d'entre eux ont le sentiment que leur situation s'est dégradée et qu'ils sont injustement pénalisés. Chez les retraités, ce chiffre atteint du jamais vu : 94 %. Et ils se sentent, de surcroît, méprisés, traités de « Gaulois réfractaires » ou de « fainéants ». Les classes populaires et moyennes sont accablées par l'impôt : hausse de la CSG pour les retraités, hausse de la fiscalité énergétique, baisse des aides au logement, si bien que la France est championne du monde des impôts et des taxes ! Ce matraquage n'est plus compris, d'autant qu'il est inefficace, puisque la dette publique continue de s'envoler, sans créer d'amélioration. Les territoires sont abandonnés, désertés par les services publics et de santé, les commerces et les transports. Et ensuite, on explique qu'il nous faut renoncer à la voiture, on surtaxe le carburant, on parsème les routes de radars qui ont généré près de 2 milliards d'euros de recettes en 2017. Vous étranglez financièrement les collectivités à coups de réductions des dotations, faisant porter sur les maires la responsabilité d'arbitrer des hausses de fiscalité. Vous êtes durs avec les Français ! La voilà la réalité. Votre politique est injuste et illisible. Pis, elle déconsidère, aux yeux des gens, la parole politique elle-même. La France qui travaille souffre : elle peine à boucler les fins de mois, elle peine à payer la cantine scolaire des enfants, elle peine à se nourrir correctement, à se loger dans le parc social, et elle peine à affronter les accidents de la vie. Depuis ce week-end, cette phrase est sur toutes les lèvres : « Les élites parlent de fin du monde, quand nous, on parle de la fin du mois. Ma question sera simple, monsieur le ministre : quand votre gouvernement va-t-il enfin passer de l'idéologie à la réalité ? Allez-vous enfin entendre la souffrance qu'expérimentent les Français, y compris ceux qui vous avaient fait confiance et qui ne croient plus en rien ? La parole

de taxes, trop de dépenses publiques et par ailleurs trop de dettes. Avouez-le avec moi- vous l'avez dit, et ce n'est pas qu'un passif récent -, de nombreux gouvernements depuis quarante ans, c'est-à-dire, permettez-moi de vous le dire, avant la naissance du Président de la République lui-même, ... ministre ! ... la France, sous diverses majorités et pour des raisons très différentes, a présenté des projets en déséquilibre. Madame la sénatrice, permettez-moi de vous dire que vous m'appelez, et à travers moi le Gouvernement, à la cohérence, c'est-à-dire à baisser les impôts. J'y suis très favorable, et pour cela, il faut baisser la dépense publique. Et j'y suis très favorable.

J'ai suivi, madame la sénatrice, vos propositions. Qu'a proposé la majorité sénatoriale ? Moins d'impôts ? Non ! Vous avez proposé de taxer les complémentaires. Non ! Ce n'est pas vrai. Si ! Vous avez proposé d'augmenter de 600 millions d'euros

Je rappelle que vous disposez de deux minutes, réplique comprise. Merci, monsieur le président. Samedi dernier, plus de 50 000 personnes se sont réunies dans toute la France pour dire « stop » aux violences sexistes et sexuelles, qui tuent une femme tous les trois jours dans notre pays. Les « féminicides » tuent, les violences conjugales blessent les femmes et, ne l'oublions pas, les enfants aussi, aspirés dans cette spirale. Nous en sommes aujourd'hui au cinquième plan de lutte contre les violences faites aux femmes. Concernant les violences conjugales, la mise en sécurité des femmes se concrétise par l'hébergement et l'accompagnement des victimes et de leurs enfants, qui doivent quitter le domicile conjugal. ces missions sont aujourd'hui remises en cause par les trop faibles moyens, les associations ont tiré les sonnettes d'alarme, la saturation des dispositifs de maraude auprès des femmes, la saturation du 115 et des centres d'hébergement de réinsertion sociale, les CHRS. La mise en sécurité inconditionnelle, immédiate et continue n'est pas assurée. Cette situation affaiblit les engagements du Président de la République qui, en novembre dernier, déclarait grande cause nationale les luttes contre les violences faites aux femmes. Madame la secrétaire d'État, pouvez-vous nous affirmer que le budget dédié à l'hébergement va être sanctuarisé en 2019 ?

d'abord rappeler que le budget du programme 137 du budget de l'État, celui qui est consacré aux droits des femmes, a été cette année pour la première fois, exécuté à 100 %. Je n'y suis pas pour rien, évidemment, mais je crois que nous pouvons collectivement remercier le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin

1 million d'euros pour les partenaires sociaux et les associations qui portent des projets contre les violences sexistes et sexuelles au travail. Le Premier ministre, Édouard Philippe, a lancé et financé depuis Matignon, une grande campagne, dotée de 4 millions d'euros, pour interpeller les témoins de ces violences sexistes et sexuelles. En 2019, c'est 530 millions d'euros que l'État consacrera à l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est un record historique ! En 2018, nous avons augmenté considérablement un certain nombre de budgets d'associations comme le Mouvement du Nid qui accompagne des personnes prostituées- plus 150 000 euros pour un budget qui a été doublé -, le Collectif féministe contre le viol- plus 60 000 euros et ensuite plus 100 000 euros -, le planning familial- plus 100 000 euros, c'est plus de 40 % -, Excision, parlons-en !- plus 300 % pour accompagner un plan voulu par le Premier ministre en vue de lutter contre l'excision -, la Fédération GAMS- budget multiplié par Toutes les subventions nationales pour les associations qui luttent contre les violences sexistes et sexuelles sont soit maintenues, soit augmentées. En moyenne, c'est plus 21,3 % d'augmentation en faveur de ces associations, y compris le 39 19- plus 120 000 euros -, etc.

... La parole est à M. Stéphane Ravier, pour la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe.

près de 183 immeubles ont été évacués pour un total de 1 377 personnes. Ce drame a mis en lumière de graves carences quant au traitement de l'habitat indigne par la deuxième ville de France, au point qu'une information judiciaire pour homicide involontaire a été ouverte. Quant à moi, j'ai déposé une demande de création d'une commission d'enquête parlementaire, ... Nous voilà bien ! ... visant à déterminer si la ville de Marseille, les adjoints ou encore l'administration ont volontairement négligé la gestion de l'habitat indigne. Rappelons que seulement dix agents de la mairie traitaient cette question Aujourd'hui, le peuple marseillais en colère demande des comptes. Si celui qui est assis au sommet de la pyramide municipale depuis vingt-trois ans apparaît comme le grand responsable de la situation, il ne saurait être le seul un sommet repose toujours sur une base. Un maire se repose sur ses adjoints. De l'ancien premier adjoint, devenu président de la région PACA, à l'ancienne adjointe à la qualité de la ville, devenue présidente de la métropole, tous les amis de vingt-trois ans abandonnent celui à qui ils doivent pourtant tout. Pendant ce temps, ce sont plus de 1 000 hommes, femmes et enfants qui sont ballotés d'un hôtel excentré à une cantine du centre-ville, sans qu'aucune information sur leur avenir

peut-être l'annonce de cet audit n'est-elle qu'un de plus, de la part d'un ministre passé maître en la matière ! Que pouvez-vous faire pour les commerçants et artisans qui ne bénéficient d'aucun dispositif pour pallier la cessation de leur activité ? L'État ne pourrait-il pas engager des négociations avec les banques et les assureurs en vue de permettre la suspension des obligations civiles au paiement d'échéances de remboursements d'emprunt, de loyers ou encore d'assurances ? Avoir passé une semaine de vacances dans le quartier le plus huppé de la ville, fait son jogging sur les plages du Prado avec le maillot de l'Olympique de Marseille sur le dos n'a apporté aucune amélioration à la vie quotidienne des Marseillais. Alors, plutôt que de courir, quand allez-vous agir à point en faveur de la deuxième ville de France ?

Vous le savez, une enquête est en cours pour déterminer les circonstances qui ont conduit au drame, ainsi que les responsabilités. Dès la survenance de la catastrophe, l'État, en association avec les autorités municipales et métropolitaines, a organisé l'expertise et la sécurisation des immeubles situés autour des bâtiments effondrés. D'autres immeubles ont été évacués par précaution et continuent de l'être. de l'être. Les personnes évacuées sont, en majorité, relogées par les services de la ville ; les autres ont été accueillies par leur famille. Dans les jours qui ont suivi, je me suis entretenue avec le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, et la présidente de la métropole, Martine Vassal. En outre, l'État a dépêché une équipe technique pour appuyer et renforcer l'expertise locale. Nous avons bien sûr

D'autres mesures permettent de s'attaquer plus fortement, notamment, aux marchands de sommeil, et un plan d'intervention en faveur des copropriétés dégradées a été lancé par Julien Denormandie.

Cet amendement vise à inscrire dans le code général des impôts une exonération complète et permanente des primes versées par l'État aux athlètes français ayant obtenu un titre olympique ou paralympique.

appliqué aux frais de transport automobile des contribuables optant pour la prise en compte des frais réels professionnels et, de manière plus générale, le plafonnement de ces derniers.

d'impôt, et certaines dépenses ne sont seulement pas chiffrées. Permettez-moi de donner quelques exemples : nous ne connaissons pas le coût du régime d'imposition séparée des plus-values ; nous ne connaissons pas le coût budgétaire du dispositif Malraux ; nous ignorons l'impact réel des déficits fonciers sur le rendement de l'impôt sur le revenu ; nous n'avons guère d'indications sur le coût fiscal réel des contrats d'assurance-vie ou des plans d'épargne. Au-delà de ces questions, nous l'avons dit, l'objectif est affiché dans un contexte de retenue à la source et d'individualisation grandissante de l'impôt, le quotient familial est appelé à se réduire peu à peu, jusqu'à s'éteindre, parce qu'il coûterait trop cher.

de la dette sociale, la CRDS, ce qui en fait une base pour le moins solide. Le second étage- l'impôt sur le revenu lui-même -est censé frapper de manière progressive et équitable les contribuables à raison de leurs ressources,

des associations dans le secteur social, dans le domaine de la santé, de l'éducation ou encore de la recherche. Chacun se félicite d'ailleurs de cette générosité, que nous encourageons par des déductions fiscales.

Ainsi, l'Institut Pasteur, fondation reconnue d'utilité publique, prévoit une baisse de 1 million d'euros de collecte auprès de ses donateurs fidèles qui, pour près de 90 % d'entre eux, sont des retraités dont le montant moyen du don est de 40 euros. La fondation Apprentis d'Auteuil, mais également l'AFM-Téléthon et l'Institut Curie, dont 25 % de la recherche est financée par la générosité des particuliers, anticipent une diminution des dons. Afin d'inciter les donateurs à confirmer leur engagement, il est proposé d'augmenter le montant de la réduction d'impôt sur le revenu accordée au titre des dons faits par les particuliers à un organisme d'intérêt général ou reconnu d'utilité publique de 66 % à 70 %, dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Le scrutin est ouvert.

Historiquement, le taux de cet abattement, qui a remplacé l'avoir fiscal, pouvait se justifier, le taux de l'impôt sur les sociétés étant de l'ordre de 50 %. Seulement, le

l'impôt sur les sociétés est tellement dénaturé par les dérogations, régimes particuliers et exemptions d'assiette qu'il est aujourd'hui avéré que son rendement est inférieur aux sommes mobilisées pour en alléger le poids sur la comptabilité des entreprises entreprises ... En pratique, on constate qu'il est très faible pour les grandes entreprises, qui jouent habilement des niches fiscales et des dérogations, et plus élevé, hélas, pour les petites entreprises, qui ne peuvent quasiment rien « optimiser »- je mets évidemment ce verbe entre guillemets. De fait, les bénéfices substantiels échappent à cette imposition grâce à divers dispositifs, notamment celui que nous appelons la « niche Copé ». Mais le summum est sans doute atteint avec le régime des sociétés mères et celui d'intégration fiscale, dont le coût excédera le rendement de l'impôt

nous vous invitons donc à suivre cette juste préconisation du Conseil des prélèvements obligatoires en soutenant notre amendement ! Quel

d'État. Le présent amendement tend à supprimer l'article 2 qui permet aux propriétaires mettant gratuitement un logement à la disposition d'une association reconnue d'utilité publique qui réalise des actions en faveur de l'accueil et du logement des personnes défavorisées de déduire le montant de la taxe foncière correspondante de leur impôt sur le revenu. Cette mesure, qui se cumulerait avec les avantages fiscaux déjà octroyés à raison de la mise à disposition à titre gratuit d'un local au profit d'un organisme d'intérêt général, constituerait un pur effet d'aubaine pour ces propriétaires. En effet, il est déjà admis que la mise à disposition à titre gratuit d'un local, lorsqu'elle est prévue dans le cadre d'un contrat de location, ouvre droit à la réduction d'impôt au titre des dons réalisés par les particuliers pour un montant équivalent au loyer que le propriétaire renonce à percevoir. le loyer que le propriétaire renonce à percevoir reste soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, desquels peut être déduite la taxe foncière. Il n'y a donc pas lieu de permettre que la taxe foncière, déjà déductible du revenu foncier, qui, de surcroît, ouvre lui-même droit à une réduction d'impôt au titre des dons, puisse être, en plus, déduite de l'impôt sur le revenu.

ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'État dans le département et destinées aux personnes [en difficulté] sont exonérés de taxe foncière sur les

au titre de la permanence des soins par les médecins libéraux installés dans des zones identifiées comme sous-dotées par les agences régionales de santé. Ce dispositif est régi par l'article 151 du code général des impôts : « La rémunération perçue au titre de la permanence des soins exercée en application de l'article de la santé publique par les médecins ou leurs remplaçants installés dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, définie en application de l'article L. 1434-4 du même code, est exonérée de l'impôt sur le revenu à hauteur jours de permanence par an. » Si cette disposition s'applique en principe aux seuls médecins installés dans des zones déficitaires et qui participent à la permanence des soins, la direction générale des finances publiques a admis dans son instruction fiscale que la condition d'exercice dans une zone déficitaire est remplie dès lors que le secteur pour lequel le médecin est inscrit au tableau de permanence comprend au moins une zone sous-dotée. Concrètement, cela conduit à une différence de traitement entre les médecins chargés de la régulation dans un département comprenant au moins une zone sous-dotée et les médecins de garde qui interviennent au niveau d'un territoire infradépartemental, nécessairement plus restreint que celui de leurs collègues régulateurs. Aussi, il convient de revenir sur cette différence de traitement en étendant expressément l'exonération prévue à l'ensemble du territoire. Cette extension contribuerait, face à l'érosion du volontariat pour effectuer des gardes, à renforcer l'attractivité de la permanence des soins ambulatoires. Quel est l'avis de la

Lorsque l'on veut que des jeunes remplacent les médecins généralistes sur le territoire, le problème se pose de la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. Bien souvent, on trouve des remplaçants qui ne veulent pas entrer dans les systèmes de garde.

où une telle démarche était mise en oeuvre depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Or les impératifs avancés pour justifier le moindre taux de crédit d'impôt appliqué à certains investissements réalisés dans le cadre de ces opérations complexes- moindre performance au regard du coût avancé -ne résistent pas longtemps, il faut bien l'admettre, face à une réalité budgétaire plus prosaïque. Car enfin, mes chers collègues, faut-il penser que le lobbying intensif des producteurs de biocarburants est plus efficace que celui des entreprises de second oeuvre du bâtiment, pour que l'on préfère continuer de perdre des recettes de TICPE à raison de l'adjonction d'huile de palme ou de soja dans le gazole plutôt que de subventionner les doubles vitrages ou les chaudières au fioul à haute performance Vous voyez bien que le caractère pour le moins incertain et mouvementé de la fiscalité ou, ici, de la non-fiscalité écologique exige manifestement que l'on fasse preuve d'un peu de recul et de réflexion.

pour mener la transition, même si ce type de crédit d'impôt peut avoir un évident effet de levier sur la réalisation effective des travaux d'amélioration des performances thermiques des immeubles. La transformation du CITE en subventions directes, que d'aucuns ont d'ores et déjà annoncée, n'est plus forcément

je suis obligé de constater que, en effet, la situation est paradoxale au lendemain du départ d'un régiment professionnel dont nombre d'officiers, sous-officiers et soldats habitaient à l'extérieur des quartiers ou des casernes.

Sans bien connaître le sujet, je trouve qu'il n'est pas complètement inutile de maintenir le bénéfice de ce dispositif. C'est la raison pour laquelle, monsieur le rapporteur général, je ne suis pas tout à fait enthousiaste à l'idée de vous soutenir, une fois n'est pas coutume

voient leur marché de l'immobilier se détériorer, y compris, au-delà de la question de l'offre, en termes de capacité pour les investisseurs à atteindre un équilibre économique sur leurs opérations, du fait de la baisse des loyers consécutive à la perte de population. Or le dispositif que nous proposons vise aussi à permettre à des investisseurs, y compris dans le cadre de la production de logements sur des terrains libérés ou après destruction de bâtiments militaires, d'atteindre plus facilement un équilibre économique sur leurs opérations dans ces communes. Ainsi, monsieur Raynal, il ne s'agit pas

car c'est déjà fait. On veut ici étendre la mesure aux communes qui se trouvent à proximité de ce périmètre ou qui ont été concernées au cours des huit années passées.

encourage la générosité des Français qui décident d'héberger gratuitement des réfugiés statutaires. Que prévoit cette disposition ? Lorsqu'un particulier accepte d'héberger un réfugié statutaire pendant quelques mois, il peut bénéficier d'un crédit d'impôt de 5 euros par nuit,

parallèlement au projet de loi Asile et immigration par le député du groupe La République En Marche Aurélien Taché, qui avait identifié toutes les mesures permettant une meilleure intégration des réfugiés statutaires dans notre pays. Il faut le savoir, un réfugié met environ dix-huit

à confirmer ce dispositif.

Nous considérons, d'une part, que l'outil fiscal n'est pas le plus adapté pour favoriser la générosité en termes d'accueil et, d'autre part, eu égard aux montants visés et à la difficulté de vérifier et de constater l'effectivité de l'accueil, que ce dispositif serait extrêmement difficile à mettre en place. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement souhaite la suppression

Gouvernement. Depuis des années, je demande à la commission des finances, comme au Sénat, qu'on accroisse la capacité d'intégration. Or, depuis des années, je n'obtiens pas un centime.

constitue une économie budgétaire importante au regard du coût de l'hébergement dans des structures publiques. Ensuite, en termes pratiques, les structures publiques sont aujourd'hui insuffisantes, et elles ne seront pas suffisantes à court terme. Enfin, en termes d'intégration, chacun le sait, l'accueil dans des familles sur le territoire est la garantie la plus efficace d'une intégration rapide et réussie. Ce n'est pas

de retirer son amendement et d'accepter cette disposition tout à fait intéressante, même si elle reste très limitée dans son ampleur,

de bénéficier d'une réduction d'impôt au titre des dépenses que représentent les cotisations aux assurances de base que celle-ci propose aux contribuables ne disposant pas de droits ouverts auprès d'un régime de sécurité sociale en France. Autrement dit, l'ensemble des cotisations payées durant l'année fiscale à la CFE pour une ouverture de droits aux assurances de base pour le cotisant et ses ayants droit seront déductibles de l'impôt.

par des contribuables résidant dans une zone dangereuse- les zones oranges et rouges -, déconseillée aux voyageurs, définie par arrêté du ministre des affaires étrangères, pour l'application de divers prélèvements fiscaux tels que l'impôt sur le revenu des personnes physiques, y compris sur les plus-values immobilières de cession à titre onéreux, la taxe d'habitation, les droits de mutation à titre gratuit et les prélèvements sociaux.

Or le changement climatique accroît considérablement les risques d'incendie, dont les coûts économiques, sociaux et environnementaux ne sont plus à démontrer. Les forêts françaises constituent des réservoirs de biodiversité et sont, à ce titre, fréquemment intégrées au sein des schémas régionaux de cohérence écologique. Les ASA de DFCI jouent donc un rôle prépondérant en matière de protection du massif pour la sécurité des biens et des personnes et pour la sauvegarde de l'emploi et de l'intégrité du territoire, ce qui constitue autant d'économies réalisées pour les communes, les départements et l'État. je vous propose tout naturellement de porter la réduction d'impôt au montant total de la cotisation versée aux ASA de DFCI jusqu'à 500 euros. Au-delà, la réduction d'impôt est plafonnée à 50 % de la cotisation, dans la limite de 1 000 euros par foyer fiscal, comme le prévoit actuellement le code général des impôts.

de 50 %. Par ailleurs, je souhaite préciser que la loi prévoit déjà un certain nombre de dispositifs d'allégement de la charge des contribuables auxquels la loi fait obligation de procéder à un débroussaillement : les dépenses engagées par les bailleurs pour la réalisation de travaux de débroussaillement des immeubles qu'ils donnent en location sont considérées comme des dépenses d'entretien intégralement déductibles des revenus fonciers. L'avantage fiscal accordé au titre de l'emploi d'un salarié à domicile s'applique aux sommes versées pour des travaux de débroussaillement

Comme nous sommes opposés à la mise en oeuvre de la retenue à la source, nous ne pouvons qu'être opposés à l'adoption des dispositions retracées dans cet article. Le prélèvement à la source semble en effet tellement simplificateur du droit fiscal qu'il faut prévoir un article relativement interminable pour adapter la situation à la nouvelle donne. Il faut notamment trouver quoi faire pour tenir compte des réductions et crédits d'impôt, notamment pour ce qui concerne les dons aux oeuvres, les frais de garde des enfants et que sais-je encore La lecture de l'article 3 montre à l'envi que d'autres voies étaient possibles pour réformer les modalités de perception de l'impôt. Mais on sait très bien que là n'est pas l'objet final de la révision de notre système fiscal et social. fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG, la sortie du champ fiscal de la sphère de la production, voilà l'objet obscur du désir des réformateurs aujourd'hui à l'oeuvre. Loin de l'égalité républicaine ! Je ne peux donc que vous soumettre l'adoption de cet amendement.

Ne pas le faire conduirait à réduire le niveau des investissements outre-mer ou à renchérir le coût de ces investissements. Dans les deux cas, les économies s'en trouveraient déséquilibrées. Je le dis avec d'autant plus de force que nombreux sont mes collègues qui savent que je ne suis pas un prosélyte de la défiscalisation et que je ne l'encourage que si je la juge nécessaire. En l'occurrence, il me semble qu'elle l'est encore pour les économies ultramarines et qu'il convient de maintenir la stabilité de son cadre légal.

il en découlera une raréfaction de l'argent, donc de l'investissement et du financement du logement social et de l'investissement productif. C'est la raison pour laquelle il faudrait réintégrer dans le mécanisme de l'acompte ces crédits d'impôt en faveur des particuliers et des entreprises.

qui vise à intégrer le crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique dans la liste des réductions et crédits d'impôt faisant l'objet du versement d'un acompte de 60 % au 1janvier 2019. Concrètement, l'intégration de ce dispositif dans le périmètre de l'article 3 permettra une facilité de trésorerie pour les exploitations de la filière de l'agriculture biologique.

ils visent des dispositifs concernant également des entreprises ou profitant à des personnes n'ayant pas de problèmes de trésorerie particuliers, comme la réduction d'impôts pour l'investissement productif outre-mer ou la réduction d'impôt pour les investissements dans le secteur du logement social ultramarin. Je précise, monsieur Lurel, que

monsieur le rapporteur

pour calculer l'avance de 60 % qui sera versée aux contribuables au 15 janvier prochain, à prendre en compte les crédits et réductions d'impôt liés à des dépenses effectuées en 2017, partant du principe

il s'agit du prélèvement à la source pour les particuliers employeurs. Vous le savez, il a été reporté au 1janvier 2020, pour l'ensemble des 3,6 millions de particuliers employeurs utilisant notamment le chèque emploi

et les particuliers employeurs de ce secteur. Il est donc prêt à passer, dès le 1janvier 2019, au prélèvement à la source pour la catégorie d'entreprises qu'il gère. Il y aurait un risque de confusion si le GUSO, à l'égard des mêmes intermittents du spectacle et des mêmes salariés,

promu notamment en matière fiscale par la loi pour un État au service d'une société de confiance. Il est ainsi proposé qu'à compter du 1janvier 2019 et pour l'année suivante les chefs d'entreprise qui emploient moins de 21 salariés ne soient pas redevables, en cas d'erreur commise de bonne foi concernant l'obligation d'effectuer la retenue à la source, des pénalités prévues à l'article 1759-0-A du code général des impôts.

les agents des collectivités territoriales qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis, dans ce pays, à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus. C'est un cas que l'on rencontre fréquemment en Belgique. Contrairement aux agents de l'État en poste à l'étranger, ces personnes sont, sauf rares exceptions, considérées comme fiscalement domiciliées à l'étranger, alors qu'un fonctionnaire de l'État est prélevé à la source en France. Partant, elles ne sont pas imposées dans les mêmes conditions que les agents publics en service en France. Leurs revenus de source française sont ainsi soumis au barème de l'impôt sur le revenu, avec un taux minimum de 20 %. De plus, elles ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu global. Nous proposons de mettre fin à cette différence de traitement. Aucune norme supra-législative ne s'oppose à ce que des agents de l'État et des collectivités territoriales en poste à l'étranger soient mis sur un pied d'égalité.

et exerçant leur activité à l'étranger en cette qualité. Les agents des collectivités territoriales et des établissements publics en sont exclus, comme le précise la doctrine administrative. Pour ce qui concerne les agents des collectivités territoriales expatriés, ils demeurent domiciliés fiscalement en France s'ils répondent aux conditions de droit commun applicables à tous les salariés expatriés. Durant leur expatriation, ils conservent leur domicile fiscal s'ils ont en France leur foyer, c'est-à-dire leurs centres d'intérêt familiaux ou le centre de leurs intérêts économiques. Ces règles s'appliquent sous réserve des dispositions des conventions internationales. Si, en application du 1 de l'article 4 B du code général des impôts, les agents des collectivités territoriales ne peuvent être personnellement considérés comme ayant leur domicile fiscal en France, ils sont imposés dans les conditions prévues à l'article 197 A du code général des impôts, avec application d'un taux minimum d'imposition. Cependant, lorsqu'ils peuvent justifier que le taux moyen d'imposition résultant du barème français appliqué à l'ensemble de leurs revenus mondiaux est inférieur à ces taux minima, le taux moyen est alors appliqué au revenu net imposable. En pratique, le contribuable établi dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'Espace économique européen lié à la France par une convention fiscale peut bénéficier du dispositif du taux moyen, en annexant une déclaration sur l'honneur,

L'incitation consiste à les faire bénéficier d'un régime fiscal favorable, en exonérant d'impôt sur le revenu la part de rémunération correspondant à la prime d'impatriation et aux activités exercées à l'étranger. Ainsi, il est proposé d'étendre aux chercheurs le bénéfice de l'exonération de l'impôt sur le revenu actuellement applicable aux seuls salariés et dirigeants de sociétés et prévue à l'article 155 B du code général des impôts. L'exonération ne vaudrait que pour l'exercice d'activités de recherche exclusivement. Par ailleurs, la rémunération de base, hors prime, demeurerait imposable. étrangers sont trop faiblement représentés en France, cette mesure pourrait concerner en rythme de croisière jusqu'à 120 chercheurs étrangers. Considérant une rémunération de base d'un directeur de recherche majorée d'une prime d'impatriation, l'exonération représenterait ainsi